L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d'un parcours qui nous a permis de trouver un accord entre députés et sénateurs, réunis au sein de la commission mixte paritaire. Je veux m'en réjouir. Cet accord repose sur des fondements solides. Vous avez permis que nous l'obtenions, madame la ministre, en annonçant fermement les dates des 13 et 20 juin, qui ne figurent pas dans le projet de loi, pour l'organisation des élections départementales et régionales. C'était important pour nous, de même qu'il était important d'avoir la garantie qu'il serait demandé au conseil scientifique, le 1 avril prochain, de se prononcer non pas sur l'opportunité de tenir ou pas les élections départementales et régionales en juin, mais seulement sur les conditions dans lesquelles la sécurité du scrutin pourrait être améliorée, ce qui fera l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement. Nous sommes heureux que vous ayez accepté le système de la double procuration et les dispositions que nous avions prises sur la prise en charge des matériels et équipements nécessaires à la sécurité du scrutin de juin prochain. Nous avons également adopté des dispositions qui concernent les machines à voter.

s'est inquiété des sources d'insécurité dans la mesure du vote que pouvait comporter l'utilisation de ces machines.

ce qui ajoute encore à la préoccupation qu'avait pu exprimer, à propos de l'élection présidentielle de 2007, le Conseil constitutionnel. l'initiative de la majorité à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté dans notre texte, que les sénateurs membres de la commission mixte paritaire ont accepté. Que prévoit-il ? Un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement dans les six mois pour envisager les conditions du recours aux machines à voter. C'est dire si votre majorité à l'Assemblée nationale considère, comme nous-mêmes, d'ailleurs, que l'utilisation de ces dispositifs ne va pas de soi et que l'alerte donnée, voilà maintenant plus de dix ans, par le Conseil constitutionnel est pleinement justifiée. avez certainement anticipé la suite de mon propos, ce qui ne me dispense pas de le tenir. Ce matin, nous avons été stupéfaits

pas pour une petite élection, mais pour l'élection présidentielle, mère de toutes les élections, on puisse, d'une part, étendre le recours aux machines à voter et, d'autre part, le faire alors que la campagne présidentielle ne serait pas achevée, c'est-à-dire, avant le dimanche du premier tour, un jour de la semaine que le Gouvernement pourrait choisir par la voie d'un décret.

des règles minimales du débat parlementaire, de la délibération, de la concertation, de la réflexion, a beaucoup surpris. Nous en arrivons à nous demander comment on peut envisager un seul instant de recourir à une expérimentation aussi hasardeuse

le dispositif technique est pour le moins surprenant ; il est également lacunaire, et il questionne la constitutionnalité de cette initiative. initiative. Il inquiète en raison des difficultés de conservation des votes, qui seront stockés pendant plusieurs jours, et ce dans une centaine de grandes villes. Oui, cela concerne non pas quelques citoyens français, mais des millions de nos concitoyens ! On s'interroge sur les risques de double vote entre la machine à voter, par exemple le mercredi, et le vote du dimanche, ainsi que sur l'impossibilité d'un recomptage manuel dans les bureaux de vote. On s'interroge aussi sur la sincérité d'un vote, qui ne pourrait pas, par hypothèse, être modifié entre ce mercredi ou ce jeudi et le dimanche, alors que la campagne continuerait et que des événements majeurs pourraient advenir, des événements le sens du vote pour les électeurs qui, avant la fin de la campagne, auraient bénéficié de cette facilité. Quelles peuvent bien être les motivations réelles d'un tel amendement ? Est-ce que, véritablement, la motivation consistant à permettre aux familles de partir en week-end et de voter quand même est satisfaisante pour la démocratie, s'agissant d'une élection qui a toujours donné lieu à une très forte participation, et ce à juste titre

La situation sanitaire, vous le savez, questionne les modalités d'exercice de notre démocratie. Nos débats, dans votre hémicycle comme à l'Assemblée nationale, ont permis de compléter utilement le texte proposé par le Gouvernement. Nous donnons ainsi à nos concitoyens des garanties qui leur permettront de choisir en toute sécurité leurs représentants dans les conseils départementaux et les conseils régionaux. Je remercie le Parlement de la qualité des travaux qui ont ainsi été réalisés. Les débats, comme le travail réalisé dans les commissions et en commission mixte paritaire, ont permis d'aboutir à un texte opérationnel et à la hauteur de l'enjeu démocratique que représentent ces deux élections importantes. La commission mixte paritaire a finalisé un texte qui tient compte des apports des deux chambres. Plusieurs mesures, auxquelles le Parlement tenait tout particulièrement, vont ainsi concourir à la bonne tenue du double scrutin de juin prochain. Il s'agit tout d'abord de bien éclairer le Parlement par un rapport, qui sera remis au plus tard le 1 avril prochain par le Gouvernement. Il portera sur la situation sanitaire et les conditions dans lesquelles le scrutin pourra se tenir. Je rappelle, à cet égard, qu'il n'y a pas de clause de revoyure automatique dans le projet de loi. Cette question a été soulevée plusieurs fois dans les débats : s'il fallait décaler de nouveau le scrutin, ce que, je le répète, le Gouvernement ne souhaite pas, il faudrait que le Parlement vote une nouvelle loi. Nous avons également été attentifs aux demandes exprimées par le Sénat et l'Assemblée nationale sur la possibilité pour les citoyens qui souhaiteront voter par procuration de pouvoir en confier deux à un même mandataire. Le Gouvernement s'est rangé à l'avis du Parlement sur ce point, dès lors que cette mesure reste limitée aux seuls scrutins locaux de juin prochain et motivée par le contexte épidémique que nous connaissons. Le Gouvernement a aussi soutenu la mesure de l'Assemblée nationale sur les numéros verts. Sera donc autorisé pour ce double scrutin l'accès des électeurs à un numéro vert gratuit, aux frais du candidat, qui pourra par ce biais, s'il le souhaite, répondre à leurs questions. De plus, plusieurs De plus, plusieurs mesures souhaitées par le Parlement permettront de faciliter la participation à la vie démocratique des candidats. Je pense, par exemple, à la publication d'un guide du mandataire financier, ou encore au report de la date limite de dépôt des comptes de campagne. Enfin, le Gouvernement s'est rangé à l'avis des deux chambres sur la date de fin de mandat pour les conseillers régionaux qui seront élus en juin prochain. Cette fin de mandat sera donc fixée à mars 2028,

la semaine dernière : les élections départementales et régionales se tiendront bien les 13 et 20 juin prochain. Ce sont les dates que le Sénat demandait. Dès la promulgation de la loi que nous examinons aujourd'hui en lecture définitive, le texte de convocation des électeurs sera signé

Le deuxième engagement pris par le Gouvernement est de faciliter l'organisation de ce double scrutin, dans le contexte particulier que nous connaissons en ce moment. Lors du débat de ce texte au Sénat, nombre d'entre vous ont insisté sur la fourniture d'équipements de sécurité. L'État l'avait déjà fait pour les élections municipales ; il est bien prévu qu'il fournisse aux communes- à ses frais, bien sûr -tous les équipements nécessaires pour organiser le double scrutin dans les conditions sanitaires les plus satisfaisantes possible. Je vous avais également indiqué que plusieurs mesures réglementaires étaient prévues pour mutualiser certaines fonctions dans les bureaux de vote. Je crois que nous avons ainsi pu répondre à une attente forte exprimée par le Parlement, qui s'était

À l'Assemblée nationale comme au Sénat, de nombreux amendements ont été déposés sur les questions relatives au vote électronique, aux machines à voter, ou encore au vote anticipé ; plusieurs appels ont été lancés par des parlementaires à cette occasion.

notamment quant à l'identité de la personne qui vote. Néanmoins, le Gouvernement a entendu cet appel. Nous travaillons à répondre à cette attente de modalités nouvelles d'expression du suffrage sans mettre en risque la validité d'un scrutin. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les élections des conseils départementaux et des conseils régionaux pourront donc se dérouler les 13 et 20 juin prochain dans les meilleures conditions possible au vu de l'épidémie que nous connaissons. Ce rendez-vous démocratique majeur sera ainsi tenu. Encore une fois, nos échanges, nos débats et votre travail ont permis de compléter utilement le dispositif proposé ; je vous en remercie.

démocratique. Notre objectif n'était pas de lui imposer une obligation supplémentaire, mais bien de la renforcer dans son rôle d'information et d'éducation civique et politique, dont nous avons besoin pour faire vivre collectivement la démocratie dans notre pays.

C'est l'essentiel : la crise sanitaire que nous traversons le commande, et il aurait été dommageable pour le Parlement que nous ne trouvions pas de consensus sur ce projet de loi. Initialement, ce texte comportait quatre articles ; aujourd'hui, il en comporte quatorze. Le Sénat a très largement contribué à son enrichissement. Je pense particulièrement à la proposition sénatoriale d'un nouveau calendrier électoral permettant de revenir au droit commun plus rapidement, dès mars 2028, à la possibilité d'une double procuration, si chère à notre rapporteur Philippe Bas, à la prise en charge par l'État des équipements assurant la sécurité sanitaire de nos concitoyens lors de ces élections, à l'utilisation d'une même machine à voter pour les deux scrutins- je ne reviendrai pas sur l'utilisation d'autres machines à voter pour d'autres scrutins ... -, au délai supplémentaire octroyé aux candidats pour déposer leur compte de campagne, ou encore à l'autorisation donnée aux départements et aux régions d'adopter leur budget primitif pour 2021 et leur compte administratif pour 2020 jusqu'au 31 juillet Saluons la sagesse des deux rapporteurs et particulièrement celle de Philippe Bas, rassuré par l'engagement du Gouvernement de renoncer à l'inscription d'une date butoir dans la rédaction de l'article 1 de ce projet de loi. Concernant le fameux rapport prévu à l'article 2, la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire aboutit à un consensus plus que satisfaisant. Je me réjouis que l'amendement déposé par Alain Richard tendant à allonger à dix-neuf jours, au lieu de douze, la durée de la campagne officielle ait été repris par l'Assemblée nationale, puis par la commission mixte J'avais évoqué, en première lecture, les difficultés matérielles que pourraient rencontrer les radios publiques et France Télévisions pour la diffusion des clips de campagne pour les élections régionales. Il me faut saluer l'article 6 , dont la rédaction finale élargit aux élections régionales la proposition sénatoriale de diffuser des programmes pédagogiques sur le rôle et le fonctionnement des assemblées départementales. Je vous

le rapport au temps. Le pouvoir que le peuple concède à ses dirigeants ne l'est que. La démocratie offre un double mécanisme protecteur au peuple souverain : éviter qu'il ne soit dépossédé de sa faculté de rester maître des horloges et garantir périodiquement des élections.

la portée ne sera sans doute pas très importante ; l'augmentation de 20 % du plafond des dépenses de campagne, compte tenu de l'allongement de la période de prise en compte des dépenses électorales dans les comptes de campagne ; l'allongement d'une semaine de la durée de campagne officielle et son passage à trois semaines une communication sur le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux et régionaux, au détriment d'un mécanisme que nous aurions souhaité plus ambitieux- j'y reviendrai.

municipales ont été le péché originel : des hésitations, aucune volonté d'adaptation et l'attente d'un retour à la normale dont on savait pourtant qu'il ne serait pas rapide.

la cerise est l'article 4 , qui demande qu'un rapport sur le recours aux machines à voter soit remis au plus tard le 1 octobre 2021 ; si j'ai bien compris, cette disposition sera caduque avant même d'avoir servi.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, en tant que sénateur non inscrit, je suis particulièrement attaché à ce que notre indépendance par rapport aux partis politiques soit respectée et notamment

Le terme " divers " doit désormais être utilisé pour tous les candidats qui n'ont pas d'attache politique. » Mme le ministre avait ajouté ceci : « Nous considérons également que cette question a déjà été débattue et tranchée.

cette circulaire ministérielle du 3 février 2020 : « La nuance, quant à elle, est attribuée de manière discrétionnaire par vos services ... »- ceux du préfet à partir des grilles annexées à la présente circulaire. Il est tout à fait possible qu'elle soit différente de l'étiquette déclarée par le candidat. » On n'a donc strictement rien changé ! C'est un énorme mensonge que de dire que l'affaire a été réglée : le préfet a toujours la possibilité

Marc. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les élections régionales et départementales étaient prévues au mois de mars prochain. Ces élections locales sont une composante essentielle de la démocratie. Or la gravité du contexte sanitaire a balayé toutes nos certitudes. La persistance de l'épidémie a conduit le Gouvernement à s'interroger sur la faisabilité de l'organisation de ces scrutins. Le projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a pour objet principal de prévoir le report de ces scrutins de mars à juin 2021. Je souhaite rappeler l'importance de ces élections. Les élus qui s'y engagent permettent de faire vivre nos collectivités. Il me faut saluer ces femmes et ces hommes qui soutiennent l'entretien de nos routes, la rénovation d'un collège ou d'un lycée, ces femmes et ces hommes qui coordonnent des plans d'aide sociale à l'enfance ou aux personnes âgées, ces femmes et ces hommes qui accompagnent hôpitaux, Ehpad et entreprises. Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune de l'ensemble des dispositions restant en discussion, car le report de ces scrutins constitue une décision sensible et exceptionnelle, directement et exclusivement liée au contexte pandémique que nous traversons. Je me félicite de l'esprit d'écoute et de dialogue constructif qui a prévalu. Le projet de loi, qui comportait initialement quatre articles, a été enrichi au Sénat de plusieurs modifications et ajouts ; je suis heureux qu'un grand nombre de nos apports aient été maintenus. En effet, l'Assemblée nationale en a accepté la majorité. Je voudrais citer l'échéance fixée à mars 2028 des prochains mandats, le recours à la double procuration, ou encore l'extension du délai de dépôt des comptes de campagne. Je pense aussi à la mention spécifique des marges d'erreur dans les sondages publiés, ou encore à la mise en place d'une campagne de communication audiovisuelle institutionnelle prévue par l'article 6 , campagne que l'Assemblée nationale a d'ailleurs étendue aux élections départementales. Un esprit consensuel a permis d'aboutir au maintien des articles 8 et 9, adoptés par le Sénat, qui étendent jusqu'au 31 juillet 2021 la faculté pour les régions et les départements de voter leur budget primitif et leur compte administratif. Je suis ravi de toutes les dispositions prévues dans le projet de loi pour assurer la protection des votants, et je me réjouis que l'État fournisse lui-même aux communes, à ses frais, les équipements adaptés permettant d'assurer la sécurité sanitaire du scrutin. À cet égard, je fais confiance aux maires et à leurs équipes pour organiser au mieux ces élections, dans le respect des gestes barrières. Madame la ministre, chers collègues, les incertitudes demeurent fortes en raison de l'émergence de différents variants, qui affectent la rapidité des contaminations, et du risque de saturation des hôpitaux. Néanmoins, notre pays est parvenu à tenir des scrutins l'an dernier. Malgré les graves difficultés sanitaires, notre démocratie tient le cap. Notre groupe votera donc ce texte. La parole est à M. Guy Benarroche.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, devant l'incompréhension qui s'est exprimée face à sa gestion des temps démocratiques depuis le report des élections municipales de l'an dernier, l'exécutif a cherché à anticiper les difficultés possibles. fait appel à Jean-Louis Debré, qui a remis le 13 novembre 2020 un rapport au Premier ministre sur les modalités d'organisation et le report de la date des élections régionales et départementales. Nul besoin de rappeler combien l'incompréhension et l'incertitude des parlementaires face à des décisions unilatérales et tardives, basées sur les données fournies par un conseil instauré et choisi par l'exécutif et rendues publiques selon un calendrier aléatoire, ont pu laisser des traces. Ce texte exprime dans son article 1 l'opinion unanime des scientifiques et des formations politiques sur l'impossibilité de maintenir un scrutin en mars et le consensus formé en faveur d'un report en juin 2021 plutôt qu'à l'automne, sachant que les scientifiques interrogés pour le rapport Debré estimaient que cette saison était plus propice à une reprise de l'épidémie, sans parler du faible impact d'une campagne menée pendant les mois d'été, ou du télescopage avec la préparation budgétaire de ces collectivités.

familiales. Cet apport récent traduisait dans les faits le rite républicain d'accompagner ses proches, souvent fragiles, pour voter. La possibilité pour les citoyens de faire appel à des OPJ pour établir leur procuration en dehors des mairies et commissariats

Notre groupe s'interroge également sur la mutualisation des machines à voter pour les deux élections et surtout sur l'ouverture par l'article 4 de la possibilité

En plus de rendre public sans délai ce rapport, le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, a souhaité rappeler que notre interlocuteur doit rester le Gouvernement, qui nous remettra lui-même un rapport à partir de l'avis des scientifiques. Ce rapport devra nous indiquer comment sécuriser la mise en oeuvre des élections, y compris pour la campagne, qui pourrait être mise à mal par le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, qui a servi de base à des décrets limitant les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique à six personnes, décrets qui seront toujours en vigueur. la commission mixte paritaire ait conservé l'article 6 prévoyant une campagne d'information audiovisuelle sur les élections régionales et départementales. Restent beaucoup de questions sans réponse.

toutes ces raisons, même si le consensus d'un vote en juin nous convient, du fait de toutes nos réserves sur l'évolution de la situation sanitaire, sur la réalité d'un nécessaire dialogue entre l'exécutif et l'ensemble des mouvements politiques et sur l'existence possible d'une vraie campagne électorale,

à un bon dialogue entre le Gouvernement et les deux chambres du Parlement : l'adaptation de la durée de la campagne, la modification du délai de dépôt du compte de campagne et des délais de candidature, ou encore

Nous pouvons dire modestement que nous avons accompli un travail législatif correct, avec un effort de réponse aux défis que nous rencontrions pour l'organisation de ces

Les exemples dans les pays voisins nous le prouvent : lorsque les gestes barrières sont respectés, les électeurs n'encourent que très peu de risques à venir voter. Ce qui me préoccupe le plus est de savoir si nos concitoyens se déplaceront les 13 et 20 juin prochain. Ne nous voilons pas la face : peu d'entre eux savent que des élections vont se tenir en juin. Nous risquons, hélas ! de battre des records d'abstention au vu de ce qui s'est déjà produit lors des municipales de 2020. À l'improvisation du premier tour avait succédé une organisation plus forte du second, plus sécurisante pour les agents électoraux et les assesseurs, qui sont en première ligne lors des opérations de dépouillement. du présent texte, les membres du groupe du RDSE restent favorables à l'augmentation des plafonds de campagne, au dépôt différé des comptes de campagne ou encore aux doubles procurations.

L'ensemble de ces éléments constitue une première étape, mais je crains que cela ne soit pas suffisant, tant les préoccupations de nos concitoyens résident aujourd'hui ailleurs. Nombre d'entre eux sont préoccupés par la sortie de crise. C'est donc à nous, politiques, qu'il revient d'y répondre. Il serait trop facile de faire peser l'abstention sur les seuls électeurs

une démocratie doit être une fraternité ; sinon, c'est une imposture », déclarait Antoine de Saint-Exupéry. Ces mots justes nous renvoient directement à une notion fondamentale que nous oublions parfois à l'heure de la crise sanitaire, celle de la participation. La participation et la confiance sont les maillons essentiels de la démocratie. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'adoption en commission mixte paritaire du projet de loi visant à reporter les élections départementales et régionales. À l'heure où la pandémie de la covid-19 fait ressortir les maux les plus profonds de notre société et génère un mal-être sans précédent, nous nous devons de réaffirmer au sein de cet hémicycle, garant des libertés, les valeurs de notre démocratie représentative.

mois. Oui, l'épidémie bouleverse nos institutions, nos libertés publiques et nos échéances institutionnelles ! Nous avons largement débattu et amendé ce projet de loi, et mon groupe se félicite de l'accord de nos deux chambres, qui confirme la volonté d'une démocratie apaisée. Nous sommes réalistes face aux impératifs sanitaires et calendaires. Cela ne signifie pas pour autant que nous acceptons de mettre durablement entre parenthèses le principe constitutionnel de périodicité des scrutins. Ces élections doivent avoir lieu- et auront lieu -, non seulement pour l'équilibre de nos institutions, mais aussi pour garantir que la parole de nos concitoyens soit entendue et que notre démocratie perdure. Comme l'a dit notre rapporteur Philippe Bas, « la démocratie ne saurait être confinée ». Reporter les élections départementales et régionales au mois de juin 2021 doit permettre de préparer leur bon déroulement. Cela n'a rien d'impossible, loin de là : nombre de nos voisins européens organisent ou ont organisé des scrutins cette année. Nous avons pu l'observer en Catalogne, pas plus tard que le week-end dernier. Tout aussi près de chez nous, l'Allemagne organisera plusieurs élections régionales et nationales à partir du mois

Il nous faut vivre avec ce virus, et, si la situation perdurait, nous devrions nous adapter tant dans notre manière de faire campagne que dans notre processus de vote. Ce texte adopté en commission paritaire permettra le recours aux doubles procurations et garantira la fourniture par l'État

De plus, notre chambre haute s'est assurée de la tenue d'un double scrutin pour éviter une fragmentation de la participation et garantir à nos administrés simplicité et sécurité sanitaire.

Après plus d'un an de crise et de sacrifices, les Français méritent de renouer avec leurs droits de participation à la chose publique- au-delà d'un droit, c'est une nécessité. droit, c'est une nécessité. D'autres apports du Sénat continuent de figurer dans le projet de loi et procèdent à des ajustements bienvenus du déroulement des scrutins et du fonctionnement des collectivités. C'est par exemple le cas de l'adaptation du calendrier budgétaire des régions et des départements, intégrée par les amendements de notre collègue Catherine Di Folco, qui permet, là encore, d'ajuster nos institutions à la crise actuelle.

Avec une efficacité qui n'est plus à prouver et habilitées à recevoir un double scrutin, les machines à voter permettent de voter dans un seul et unique bureau, en minimisant les risques de contamination. Elles diminuent aussi le nombre de personnes engagées dans la gestion des bureaux de vote- point qui n'est pas négligeable en période de crise sanitaire -, permettant ainsi d'envisager une organisation simplifiée et adaptée aux plus petites communes. À l'heure où la démocratie cherche à se réinventer, le débat autour du moratoire des machines à voter prendra une place prépondérante dans les discussions que nous tiendrons

Espérons que les communes qui le souhaitent pourront rapidement se doter de machines nouvelle génération, une fois le moratoire levé. Espérons aussi que les discussions qui auront lieu jeudi prochain ne soient pas l'arbre qui cache la forêt de l'utilisation régulière et constante des machines à voter dans de nombreuses communes

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, tout engagement génère des compromis. C'est le propre même de notre système bicaméral, qui impose la conciliation des points de vue, sans renier ses convictions, pour aboutir à l'adoption de réformes conformes à l'intérêt général. C'est dans cet esprit que le Sénat a abordé l'examen

en commission mixte paritaire qui entérine des avancées attendues dans la lutte contre la délinquance des mineurs. En effet, la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 était devenue urgente. Les signaux de son épuisement sont nombreux, à commencer par des délais de jugement des mineurs délinquants trop longs, dix-neuf mois en moyenne- des mois qui durent des siècles quand on a 17 ans ... Cette lenteur ne permet plus à la justice d'apporter une réponse pénale efficace aux mineurs, souvent devenus majeurs lors de leur jugement. Le taux d'incarcération en détention provisoire de plus de 80 % des mineurs emprisonnés prouve, là aussi, la faillite de notre système pénal. Mais urgence ne veut pas dire précipitation. Certes, la réforme de la procédure pénale des mineurs est un sujet mûrement réfléchi qui a mis du temps à se réaliser. Dès 2008, le rapport Varinard proposait au garde des sceaux de l'époque l'introduction de la césure. Depuis lors, pendant dix ans, de nombreux rapports parlementaires ont alimenté la réflexion sur la lutte contre la délinquance des mineurs, tels que celui, réalisé par nos anciens collègues Catherine Troendlé et Michel Amiel, qui était relatif à la réinsertion des mineurs incarcérés.

attendue par l'ensemble des acteurs de la justice des mineurs- magistrats spécialisés, avocats, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, greffiers ... -, mais elle engage aussi la transformation de leurs pratiques professionnelles, ce qui génère de nombreuses craintes.

car nous sommes persuadés que les nouveaux outils juridiques permettront de mieux répondre à l'évolution de la délinquance des mineurs. C'est pourquoi le Sénat a, dans sa grande majorité, considéré que la césure, qui est au coeur de la réforme en ce qu'elle allie une audience de culpabilité, un temps éducatif et une audience de sanction, permettra non seulement d'accélérer la procédure, mais surtout de favoriser sa compréhension par le jeune qui en fait l'objet. L'efficacité de la réponse pénale réside dans la réactivité et la pédagogie.

notamment de l'âge du discernement. Si celui-ci fait débat, nous pensons que l'âge pivot de 13 ans est conforme au droit positif français, et nous nous réjouissons que l'introduction de la définition du discernement dans la partie législative du code pénal des mineurs ait été reprise par les députés ; elle guidera le juge dans son appréciation. revanche, nous regrettons que le principe de spécialisation des juridictions pour les mineurs ne soit pas appliqué dans son ensemble. Dès lors, le recours au juge des libertés et de la détention (JLD), même habilité, pour la mise en détention du mineur avant l'audience de culpabilité, ne nous paraît pas totalement garantir le principe de spécialisation. De De même, le maintien de la compétence du tribunal de police pour juger les mineurs auteurs de contraventions des quatre premières classes demeure une entorse au principe de spécialisation du juge des enfants, garant d'une justice plus éducative. nous entendons l'argument du Gouvernement sur les difficultés qu'engendrerait un transfert supplémentaire de contentieux dans les cabinets des juges des enfants, alors même qu'ils doivent mettre en oeuvre une réforme venant modifier leurs pratiques. La réussite de la réforme dépendra des moyens humains et matériels, notamment informatiques, qui seront affectés aux juridictions des mineurs. Elle dépendra surtout de la fluidité et de l'agilité de la nouvelle procédure, pour mieux répondre à la délinquance des mineurs. Cela imposera un renforcement des liens entre magistrats spécialisés et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, afin qu'aucun temps de latence entre les différentes étapes de la procédure ne vienne allonger le temps judiciaire et que la continuité éducative soit pleinement assurée. À cette fin, le Sénat a adopté plusieurs amendements, repris dans le texte de la commission mixte paritaire, ayant pour objet la numérisation du dossier unique de personnalité, l'obligation de fixer la date de mise en oeuvre de la prise en charge éducative par la protection judiciaire de la jeunesse à l'audience de culpabilité et la possibilité de convoquer les parents par tous moyens afin d'éviter des reports d'audience pour de simples raisons formelles.

Vous l'aurez compris, le Sénat se satisfait du texte adopté en commission mixte paritaire. Notre chambre a été entendue sur bien des aspects, en manifestant une volonté de sagesse et de détermination dont nous pouvons nous féliciter. Ce nouveau code de la justice pénale des mineurs démontre notre attachement à la protection de l'enfance, à la responsabilisation des parents, à l'efficacité de la nouvelle procédure pénale et à la clarification du droit, pour une meilleure lutte contre la délinquance des mineurs. Nous vous invitons donc à adopter ce projet de loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs ans se sont écoulés depuis le 2 février 1945. C'est tout un symbole que nous consacrons aujourd'hui : adopter un code dédié à la justice pénale des mineurs, fondé sur les valeurs de la République voulues par le général de Gaulle. Les modifications successives en avaient fait un texte devenu illisible ; il fallait donc le moderniser. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente », peut-on lire dans le préambule de l'ordonnance de 1945

et efficace. Ce code renforce la primauté de l'éducatif, tout en permettant une réponse pénale cohérente et encadrée dans des délais de procédure. En instaurant une réponse judiciaire plus proche de l'acte commis, nous rapprochons la justice de nos concitoyens. À proximité de leurs actes, les mineurs seront déclarés responsables pénalement ; avec souplesse, ils seront pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative unique modernisée. Je souhaite remercier tous les parlementaires qui viennent d'acter des accords politiques rares à l'occasion de la commission mixte paritaire conclusive, puis, cet après-midi, lors du vote du texte à l'Assemblée nationale. Je tiens, madame la rapporteure Canayer, à saluer votre travail rigoureux et constructif, ayant permis d'aboutir à un texte équilibré. Guidés par l'intérêt supérieur du mineur, nos débats ont permis de faire ressortir le consensus démocratique que nous devions collectivement à nos enfants. vous étiez convaincus de la nécessité de cette réforme. Vous étiez aussi impatients de contribuer à l'enrichissement du texte et avez pu aborder des questions essentielles en introduisant la définition Vous avez souhaité garantir l'effectivité d'une prise en charge éducative rapide, en imposant la communication au mineur d'une date de mise en place de la mesure dès la première audience. Vous avez étendu l'accès direct au dossier unique de personnalité aux professionnels du secteur associatif habilité. associatif habilité. Vous avez su dépasser les inquiétudes légitimes liées à la nécessaire évolution des pratiques professionnelles, en actant un report de l'entrée en vigueur de la réforme au 30 septembre 2021. S'ouvre alors une nouvelle étape, celle de sa mise en oeuvre. Soyez Soyez assurés que ce délai supplémentaire sera bien mis à profit pour préparer les acteurs de la justice des mineurs et faire en sorte qu'ils s'approprient ce texte,

greffiers, magistrats, avocats : tous sont engagés dans la mission si difficile de redonner de l'espoir à nos enfants. Je veux plus particulièrement remercier toutes les équipes de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est une grande direction, quotidiennement engagée dans la prise en charge des enfants, qui a fait la preuve de sa capacité normative à faire évoluer le droit des mineurs et, ainsi, toute notre société. Vous avez, durant les débats,

j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Je ne doute pas que chacun ici conserve à l'esprit les apports bienvenus de ce texte. C'est un texte nécessaire et équilibré, qui ne laisse pas le répressif prendre le pas sur l'éducatif et qui ne met pas non plus de côté l'impérative protection de notre société. Je tiens avant tout à saluer le travail réalisé tant par la commission mixte paritaire que par notre rapporteur Agnès Canayer. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont finalement réussi à se mettre d'accord sur un texte commun, grâce à un travail apaisé et constructif autour d'un sujet parfois sensible mais toujours exigeant.

merci de permettre au texte d'Annick Billon de prospérer ; merci de reconnaître que la bonne idée peut venir du Sénat ; merci de nous aider à trouver la possibilité d'obtenir ce que nous n'avions pas obtenu en 2018 de votre prédécesseure. Je salue enfin Annick Billon, qui a su tenir bon dans la tempête. Mais revenons à nos mineurs auteurs et à ce texte de compromis. Mon groupe, comme tous les professionnels qui nous avaient alertés, est satisfait du report de l'entrée en vigueur de cette réforme au 30 septembre prochain prochain ; de la précision apportée sur le discernement du mineur, question centrale de cette réforme, en lien direct avec la présomption d'irresponsabilité pénale du mineur de 13 ans

Certes, nos deux assemblées s'accordaient sur la nécessité, au nom du principe de l'impartialité du juge se prononçant sur la culpabilité, d'impliquer un autre magistrat concernant la détention provisoire. provisoire. L'Assemblée nationale a choisi le JLD, tandis que nous souhaitions confier cette mission à un autre juge des enfants, au nom de la spécialisation. Au final, c'est la position de l'Assemblée nationale qui l'emporte.

qui est la clé de voûte de la justice des mineurs, car elle porte, avec l'aide du secteur associatif habilité, l'essentiel du volet éducatif. C'est pourquoi la PJJ doit être dotée de moyens humains, financiers et matériels lui permettant d'accomplir sa mission. Son succès profitera tant aux mineurs, qui doivent avoir une réelle chance de se réinsérer, qu'à la société. L'enjeu est à cet égard bien plus grand que le texte qui nous occupe aujourd'hui.

Ces dernières années nous l'ont trop souvent douloureusement rappelé, ceux qui ont attaqué la France en son coeur étaient souvent connus des services de police pour des faits de délinquance alors qu'ils étaient mineurs, avant de basculer dans le séparatisme religieux. En rupture avec la société lorsqu'ils étaient mineurs, ils le furent avec la République et ses valeurs, une fois adultes. En définitive, la PJJ doit pouvoir exercer pleinement son rôle éducatif

Vous nous avez entendus concernant les enfants victimes, monsieur le garde des sceaux, je ne doute pas que vous nous entendrez sur la protection qu'il est indispensable d'apporter à l'ensemble des mineurs, en particulier à ceux qui se détournent du droit chemin. Vous l'aurez compris, notre groupe votera ce texte de compromis.

Premièrement, nous pensons, et cela a d'ailleurs été dit à plusieurs reprises au cours du débat, que la spécialisation de la justice des mineurs est un principe qui doit être absolument respecté. Or tel n'est pas le cas dans ce texte. Je pense à deux dispositions que vous connaissez par coeur, madame la rapporteure. Tout d'abord, la compétence du tribunal de police sa réapparition, alors que le Sénat avait jugé qu'elle était totalement contraire au principe de spécialisation. Personne ne peut dire le contraire.

Cet amendement a été supprimé en CMP. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas qui, ici, pourra défendre l'idée selon laquelle cette loi ne doit pas prendre en compte le secteur associatif habilité. Il n'y a pas de raison. Comme il n'y a pas de raison, je comprends mal la position de la CMP. Troisièmement, cette réforme ne permet pas de faire face au problème majeur du manque de moyens matériels et humains auquel sont confrontés les professionnels judiciaires et de la protection de l'enfance.

connaissez par coeur : la présomption irréfragable de non-responsabilité pénale d'un mineur de 13 ans, laquelle n'a pas été adoptée. Nous avons beaucoup argumenté

les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, [ ...], et en particulier d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale

l'ordonnance du 2 février 1945 est devenue difficilement lisible et compréhensible en raison de la sédimentation des réformes législatives fois modifié, ce texte a perdu peu à peu efficacité et cohérence. Ainsi, il ne permet plus de répondre aux exigences en matière de respect des droits de l'enfant et d'efficacité de la lutte contre la délinquance des mineurs. Aussi, l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs participe à atteindre l'objectif de modernisation de la justice pénale des mineurs. Toutefois, nous déplorons un certain manque d'ambition, un acte manqué : nous espérions un véritable « code des mineurs » réformant à la fois l'enfance délinquante et l'enfance en danger. Malheureusement, l'enfant délinquant est en effet trop souvent un enfant victime de carences éducatives ou de l'absence de parents. Réunie le 4 février dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 11 septembre 2019 a été conclusive. Je me réjouis que, grâce à des efforts conjoints, des compromis aient été trouvés permettant d'aboutir à un accord, comme cela a souvent été le cas depuis le début de la législature. À cet égard, je salue l'esprit de responsabilité et de consensus du Parlement. Je suis heureux qu'un certain nombre d'apports du Sénat aient été conservés. C'est le cas de l'introduction de la définition du discernement à l'article 1 A. C'est également le cas, à l'article 6, de la possibilité de numériser le dossier unique de personnalité, dont l'accès sera désormais autorisé au personnel du secteur associatif habilité afin de faciliter la circulation des informations entre les nombreux acteurs de la justice des mineurs. La commission mixte paritaire a aussi jugé pertinent que la date de mise en place des mesures éducatives soit communiquée au mineur à l'issue de son audience de culpabilité et a conservé la disposition visant à permettre que la convocation des représentants légaux se fasse « par tout moyen ». La CMP a également maintenu deux mesures qui protégeront nos mineurs et faciliteront leur réinsertion : l'obligation de disposer des réquisitions du parquet pour placer un mineur sous contrôle judiciaire, quel que soit le stade de la procédure, et l'effacement simplifié des dispenses de mesures éducatives et des déclarations de réussite éducative dans le casier judiciaire. Enfin, concernant l'entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, les députés, qui s'étaient montrés très attachés à la date du 31 mars 2021, se sont ralliés à la position du Sénat, qui proposait un report de six mois, au 30 septembre 2021, afin que les juridictions puissent préparer dans le calme la transition vers les nouvelles procédures. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il apparaît particulièrement nécessaire de remplacer l'ordonnance de 1945 par un ensemble cohérent de mesures susceptibles de clarifier les procédures applicables et d'apporter une réponse plus efficace aux infractions commises par les mineurs. Avant tout procédurale, cette réforme est équilibrée. Elle n'entraînera ni une moindre pénalisation ni une surpénalisation des mineurs, mais devrait permettre une meilleure organisation du procès. Notre groupe votera ce texte.

sur le présent texte, celui-ci ne convient pas au groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, au nom duquel je m'exprime devant vous. vous. Nous demandions la suppression dans le code de la justice pénale des mineurs de la mesure de retenue, pouvant aller jusqu'à douze heures, d'un jeune âgé de moins de 13 ans par un officier par un officier de police judiciaire, rappelant que la présomption d'irresponsabilité s'appliquait à ces mineurs. Nous nous sommes opposés au maintien des dispositifs de surveillance électronique en cas d'assignation à résidence, avec port du bracelet électronique, rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure adaptée aux enfants et aux adolescents, qui ne la comprennent pas. Nous demandions la suppression de l'article du code ouvrant la voie à une exception à l'excuse de minorité, estimant qu'il n'était pas concevable que le jeune âge de ces mineurs ne soit pas automatiquement pris en compte pour leur appliquer des atténuations de peine. Nous demandions également l'inscription dans ce code de l'interdiction de l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuels, soit la visioconférence, tout au long d'une procédure mettant en cause un mineur, car celle-ci contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous avions appelé de nos voeux l'instauration d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 14 ans, ce qui aurait permis à la France de se mettre en conformité avec la convention internationale des droits de l'enfant, tout en appliquant un seuil déjà retenu dans plusieurs autres pays européens. Enfin, nous avions tenté de réaffirmer la primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives en consacrant ce principe cardinal de la justice pénale des mineurs dans l'article préliminaire de ce code. Aucune de ces améliorations ne figure dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui. Nous ne pouvons que le regretter. L'ordonnance de 1945 était un texte novateur et protecteur en matière de justice des mineurs, notamment parce qu'il était fondé sur une vision bienveillante du droit face à des jeunes en pleine construction. Aujourd'hui, nous déplorons que les mesures de contrôle se substituent aux mesures éducatives, que les solutions d'insertion retenues prennent de moins en moins en compte le projet de l'enfant,

du fait du dangereux rapprochement effectué entre ce droit et le droit pénal général, qui concerne avant tout les majeurs. Ce texte ne nous satisfaisait pas en première lecture. Tel qu'il résulte des travaux de la CMP, il n'est toujours pas conforme à la vision de la

L'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, qui avait fait l'objet d'une quarantaine de modifications, contribuant chaque fois à rendre son contenu un peu plus illisible pour l'ensemble des acteurs concernés, ne permettait plus de faire face aux enjeux de la nouvelle délinquance des mineurs. Ce texte, sur lequel nous sommes parvenus à un compromis équilibré, est le fruit d'une longue réflexion sur le sujet. Entamée en 2008 par la commission Varinard, la réforme a joué l'Arlésienne jusqu'à l'ordonnance présentée le 11 septembre 2019. Le nouveau code est d'une importance majeure, car il met en place une modernisation historique de la justice pénale des mineurs afin de faire face aux enjeux de la délinquance dans notre pays, laquelle fait régulièrement la une de l'actualité, tout en conservant ses principes fondateurs : la primauté de l'éducatif, la spécialisation des juridictions et l'atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge. La nouvelle procédure de mise à l'épreuve éducative renforcera le sens de la réponse pénale, et ce dans un délai raisonnable, aussi bien pour le mineur que pour la victime, qui bénéficiera d'une réparation plus rapide. Conformément aux engagements du Gouvernement, un débat approfondi et constructif a pu s'engager au cours de la navette. Malgré les craintes initiales, et légitimes, liées au fait que la réforme se fasse par ordonnance, l'ensemble du code a pu être discuté et amendé. Et le Parlement l'a fortement enrichi ! Ainsi, l'Assemblée nationale a introduit dans la loi la référence à l'intérêt de l'enfant dès l'article préliminaire. Elle a renforcé les garanties dans le cadre de l'audition libre, interdit la visioconférence pour le placement en détention provisoire et simplifié le cumul des mesures éducatives et des peines. Le Sénat, quant à lui, a inscrit dans la loi une définition du discernement, la numérisation du dossier unique de personnalité, auquel le secteur associatif habilité pourra avoir accès, ou encore la convocation des représentants légaux par tout moyen. Les discussions se sont poursuivies lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur les quelques points de divergence qui subsistaient entre nous. Permettez-moi d'ailleurs de saluer le travail considérable des rapporteurs et la très grande qualité de nos échanges. Nous sommes parvenus à nous mettre d'accord, sans revenir sur les principes de spécialisation et d'impartialité, sur le rétablissement de la compétence du juge des libertés et de la détention en matière de placement en détention provisoire d'un mineur et sur celle du tribunal de police pour les contraventions les moins graves.

Bien sûr, la réussite de la présente réforme reposera sur les moyens mis à la disposition de la justice pénale des mineurs. La forte hausse des crédits alloués à la justice pour l'année 2021 démontre que la volonté politique est là. Mais, vous l'aurez compris, monsieur le garde des sceaux, nous serons nombreux à nous montrer vigilants quant à leur mise à disposition effective. Pour l'ensemble des raisons évoquées, le groupe RDPI votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

Il s'agissait bien sûr d'apporter une réponse pénale adaptée à l'enfance délinquante, mais avant tout d'entretenir l'esprit de l'ordonnance de 1945, qui consacre la primauté de l'éducatif sur le répressif, la spécialisation des juridictions, ainsi que l'atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge. Enfin, l'enjeu était de mieux accompagner les mineurs et de leur éviter de sombrer dans une délinquance durable. Il n'est pas commun de se satisfaire du report de l'entrée en vigueur d'une réforme, mais permettez-moi de le faire ici. Une mise en oeuvre de la réforme dès le mois prochain aurait été très compliquée et aurait donné lieu à l'application de deux procédures, qui se seraient chevauchées, comme nous l'avions indiqué en première lecture. Aussi, je me réjouis que la CMP ait pu trouver un accord sur ce point. Concernant le discernement, là encore, un pas a été fait en notre direction, la définition que nous avons introduite à l'article 1 A La fixation d'un seuil de discernement est aussi la bienvenue, car elle permet à la France de se mettre en conformité avec les accords internationaux. Le choix d'une présomption simple est difficile, mais selon moi nécessaire, afin de limiter les effets de seuil et de laisser une libre interprétation au juge. La CMP a enfin amélioré le texte à l'article 6 . Le texte prévoyait le doublement de l'amende encourue par les représentants légaux de mineurs poursuivis qui ne répondent pas à une convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs. Son maintien aurait représenté une double peine pour des familles souvent très fragiles socialement et économiquement. Son remplacement par l'obligation de participer à un stage de responsabilité parentale est en ce sens une solution équilibrée. Je ne réitérerai pas mes craintes sur l'audience unique, que je redoute de voir se généraliser, sur l'accent davantage mis sur la privation de liberté que sur les mesures éducatives ou encore sur les moyens financiers qu'il faudra continuer à mobiliser pour que cette réforme soit effective et qu'elle améliore considérablement considérablement le traitement de la jeunesse délinquante. Cette amélioration devra nécessairement passer par un recours plus faible à la détention provisoire, car l'enfermement n'est jamais une solution en soi. Il est même parfois, hélas ! le début d'un parcours carcéral continu. Pour conclure, je rappellerai les propos que j'ai tenus lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Monsieur le garde des sceaux, j'avais souhaité que nous ayons un réel débat sur un texte aussi fondateur, au vu des circonstances dans lesquelles il nous avait été présenté. Malgré la procédure accélérée et grâce au travail de nos deux assemblées- je remercie notre rapporteur Agnès Canayer pour son engagement sur ce texte -, je pense que le débat a pu être mené jusqu'au bout.

À l'issue de nos débats, au regard des conclusions de la commission mixte paritaire, un certain nombre de questions demeurent

Alors, oui, on réaffirme collectivement les grands principes, à condition, finalement, que ceux-ci n'aient pas d'effets sur la hauteur des piles de dossiers en attente. Alors, oui, on va plus vite,

projets de loi d'organisation de la justice : aller un peu plus vite, toujours plus vite, avec des effectifs réduits. Malheureusement, ce texte n'y échappe pas. le seul moyen d'accélérer les délais de jugement sans augmenter les effectifs est finalement de rogner le principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif et le principe de l'atténuation de la responsabilité du mineur. Nous proposions dans le

! Ne boudons pas notre plaisir. L'accord trouvé en commission mixte paritaire est un double succès, dont le groupe Les Républicains se félicite. D'une part, députés et sénateurs sont tombés d'accord sur le fond du texte, qui deviendra, demain, le nouveau code de justice pénale des mineurs.

Il s'agit donc d'un ralliement tardif, mais heureux, puisqu'il bénéficiera directement aux acteurs de cette justice singulière qu'est la justice pénale des mineurs. Nous le disons de nouveau : ni les magistrats ni les moyens informatiques n'étaient prêts. À l'évidence, trouver un compromis en commission mixte paritaire nécessitait de renoncer à certaines dispositions, et nous ne pouvons que regretter la disparition de deux apports du Sénat. En premier lieu, le transfert au juge des libertés et de la détention de la compétence en matière de placement en détention provisoire d'un mineur aura bien lieu. Le Sénat souhaitait que cette compétence soit confiée à un juge des enfants distinct de celui saisi, pour respecter l'impartialité, considérant que le juge des libertés et de la détention n'est pas nécessairement spécialisé en droit pénal des mineurs. En second lieu, nous nous étions opposés à ce que le tribunal de police puisse juger les mineurs pour les contraventions des quatre premières classes. Nous estimions en effet que certaines de ces contraventions sont graves pense aux violences volontaires, même si elles ne sont pas suivies d'une interruption totale de travail - et qu'elles pouvaient nécessiter un suivi éducatif particulier, afin d'éviter la récidive. À cet égard, notre collègue député Jean Terlier estimait le nombre de poursuites à l'encontre de mineurs pour des contraventions des quatre premières classes à 5 000 affaires par an. Il jugeait à ce titre que, si l'on aspirait à « alléger le travail de la justice, ce n'était pas le moment de remettre dans le circuit un volume d'affaires aussi important ». Cependant, l'on perçoit en creux que ce choix se fonde sur l'insuffisance de moyens humains.

2020, ne suffit pas, pas plus que les « sucres rapides » chers à la Chancellerie, laquelle semble désormais trouver de l'inspiration dans le travail des nutritionnistes ... Néanmoins, plusieurs apports du Sénat ont été maintenus dans le projet de loi final. Ainsi, nous saluons l'interdiction du recours à la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire d'un mineur. De même, nous nous félicitons de l'introduction de la définition « sénatoriale » du discernement - nous sommes des experts qui devait intervenir au niveau réglementaire et qui sera finalement inscrite dans la loi. Le Sénat a également souhaité rendre possible la numérisation du dossier unique de personnalité et d'y donner accès au personnel du secteur associatif habilité, ce qui facilitera sans nul doute les échanges entre les professionnels chargés de la justice des mineurs. La fluidité de la transmission des informations profite à tous, et la justice a tout à gagner quand les moyens lui sont donnés d'apporter des réponses rapides. Enfin, une autre disposition issue du Sénat permettra l'effacement simplifié des dispenses de mesure et des déclarations de réussite dans le casier judiciaire. Cet ajout nous semble particulièrement bienvenu, puisqu'il participe au relèvement éducatif et moral des mineurs, principe fondamental en matière de justice des mineurs, réaffirmé par le nouveau code de justice pénale des mineurs. Alors qu'elle a régulièrement été qualifiée de « serpent de mer », cette réforme est sur le point d'aboutir. À cet égard, nous saluons la qualité des travaux préparatoires effectués en la matière, sont issus de la mission d'information du Sénat sur la réinsertion des mineurs enfermés, menée par nos anciens collègues sénateurs Catherine Troendlé et Michel Amiel. Le groupe Les

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote

dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l'ensemble du projet de loi.